La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 17 mai 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté.

En effet, en application du premier alinéa de l'article 92 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts. Dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %. Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa de l'article 92 précité sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Il résulte de ces dispositions que les recettes tirées de la présence d'éoliennes dans les bois et forêts qui relèvent du régime forestier sont prises en compte dans l'assiette des frais de garderie.

à réaliser. Chaque forêt bénéficie ainsi d'une gestion adaptée à ses spécificités. En contrepartie de cette gestion, les collectivités territoriales doivent verser à l'Office national des forêts des frais de garderie assis sur tous les produits de leur domaine

de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. En conséquence, les recettes tirées de la présence d'éoliennes dans les bois et forêts qui relèvent du régime forestier sont prises en compte dans l'assiette des frais de garderie. Le développement de l'énergie éolienne dans les forêts peu productives offre une ressource financière complémentaire non négligeable pour les collectivités territoriales ; le Gouvernement y est très sensible. De plus, l'application du régime forestier à tous les revenus des forêts communales permet de financer les activités de l'ONF. Je rappelle que, moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'ONF des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités territoriales sont assurées sans aucuns frais par l'établissement public. Les frais de garderie contribuent à hauteur de 17 % au coût de l'application du régime forestier dans les forêts des collectivités. Le reste est financé par l'État au travers du versement compensateur attribué à l'Office national des forêts. Au regard des services rendus par l'ONF, vous comprenez qu'il n'est pas envisageable d'exclure de l'assiette des frais de garderie les recettes tirées de la présence d'éoliennes. Une telle exclusion ouvrirait la porte à d'autres demandes et serait de nature à remettre en cause l'équilibre dégagé entre l'État, les communes forestières et l'Office national des

entraîner la suppression de 38 postes d'enseignants dans les écoles rurales. Ces postes vont être redirigés vers des écoles de quartiers prioritaires. Les fermetures de classes rurales vont donc permettre de pourvoir les emplois nécessaires aux dédoublements des classes de la métropole mancelle. Les territoires ruraux sont donc bien les variables d'ajustement de votre politique éducative ! Le Gouvernement doit comprendre que nos campagnes doivent être traitées de la même manière que les zones urbaines défavorisées. Ainsi, le seuil de fermeture des classes devrait être divisé par deux en milieu rural, comme il est divisé par deux dans les zones urbaines d'éducation prioritaire. De nombreuses communes rurales de la Sarthe ont été classées en zone de revitalisation rurale, ou ZRR, ce qui revient

La base de notre pays, c'est l'école, c'est la première des batailles que j'avais définies. » Encore faudrait-il se donner les moyens de la remporter sans que l'effort se fasse au détriment des élèves des campagnes ! Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour apaiser la colère des écoles rurales ?

un meilleur taux d'encadrement sur l'ensemble du territoire dans le premier degré. Ainsi, le ratio du nombre de professeurs pour 100 élèves sera de 5,55 à la rentrée 2018, contre 5,46 à la rentrée 2017. Pour mémoire, il s'élevait à 5,20 à la rentrée 2012. Dans chaque département, il y aura donc davantage de professeurs par élève à la rentrée 2018 dans le premier degré.

aucun poste n'est supprimé dans ce département. Or, si la baisse démographique avait été répercutée de manière automatique, quarante postes auraient été supprimés. Le ratio du nombre de postes d'enseignants en équivalents progressera donc à la rentrée 2018 : il passera à 5,44, contre 5,22 en 2017. Le nombre d'élèves par classe en milieu rural restera inférieur au nombre d'élèves par classe en milieu urbain, hors éducation prioritaire. Enfin, aucune fermeture d'école n'est prévue dans ce département pour la rentrée 2018. Bien entendu, les services de l'éducation nationale sont très sensibilisés à la situation de l'école en milieu rural. La carte scolaire prévisionnelle du département de la Sarthe

les agents engagés par contrat unique d'insertion- contrat d'accompagnement dans l'emploi, ou CUI-CAE, recrutés sous contrat de droit privé et relevant donc du code du travail.

J'insiste sur le paradoxe incroyable que constitue l'obligation faite aux directeurs des établissements de recruter de nouveaux AVS pour remplacer ceux qui étaient en poste.

Il est donc urgent de changer les procédures de recrutement et de pérenniser l'emploi des AVS. Je m'interroge sur la logique du système, alors que le Gouvernement a fait de l'inclusion des personnes handicapées une véritable priorité.

Depuis la rentrée 2014, les AESH se sont substitués sur la mission AVS aux assistants d'éducation, ou AED. Ils interviennent selon les mêmes modalités que les anciens AED-AVS. Votre question porte spécifiquement sur l'enseignement privé, mais je précise

CUI-AVS. Contrairement aux AED, les AESH ont la possibilité d'accéder à un CDI, après six années d'engagement en CDD. Les candidats aux fonctions d'AESH doivent être titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne. Toutefois, peuvent être dispensées de la condition de de la condition de diplôme les personnes qui ont exercé pendant au moins deux années les fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. L'accès à un contrat d'AESH est possible pour

C'est le cas de la commune d'Aizenay, en Vendée, dont la population est passée de 6 095 à 9 212 habitants en quinze ans. Cette commune bénéficie actuellement de la DSR à hauteur de 794 000 euros.

commune perdrait donc plus de 700 000 euros de dotations, pour la simple raison qu'elle aura franchi le seuil symbolique de 10 000 habitants. Ce système de paliers est extrêmement pénalisant pour les communes. Maintenir ce seuil n'encourage d'ailleurs pas la création de communes nouvelles. En effet, un pacte financier garantit pendant trois ans le niveau des dotations de l'État aux communes fusionnant au sein de communes nouvelles de moins de 10 000 habitants, avec une majoration de 5 %.

la seconde serait d'instaurer une dégressivité sur cinq ans, par exemple, de la dotation de solidarité rurale, jusqu'à parvenir au niveau de la dotation de solidarité urbaine.

en hausse de 8,5 %- cette dotation s'élève à 1,7 million d'euros, contre 1,6 million d'euros l'année dernière. Cette augmentation résulte notamment de la progression de la dotation de solidarité rurale, qui voit son montant augmenter pour atteindre 867 000 euros en 2018. Toutefois, je je précise que le montant que cette commune devrait percevoir en 2021 ne peut être garanti. En effet, la DGF est une dotation que l'on qualifie de « vivante » : elle évolue chaque année en fonction de critères de ressources et de charges, et ne suit pas une trajectoire linéaire, commune par commune.

Un tel effet de seuil est inhérent aux mécanismes de répartition. Il est en effet indispensable de fixer des seuils au-dessus ou en dessous desquels les communes sont ou ne sont pas éligibles à tel ou tel dispositif. Si l'on ne procède pas ainsi, on dispersera nécessairement les concours financiers de l'État entre l'ensemble des collectivités. Ce n'est pas là une simple réponse théorique, il s'agit d'un cas tout à fait concret : tout élargissement de la liste des communes éligibles à une dotation réduit d'autant les montants attribués aux autres communes. Ainsi, en 2018, seize communes ont dépassé en métropole le seuil de 10 000 habitants. Si leurs

constitutionnel exige également que les seuils ne produisent pas des effets disproportionnés pour ceux qui y sont soumis. Sur ce point, vous observez vous-même que le passage au-dessus des 10 000 habitants permet souvent à une commune perdant son éligibilité à la DSR de devenir bénéficiaire de la DSU : on peut citer, par exemple, la commune de Juvignac, dans l'Hérault, qui a perdu 107 000 euros de DSR et gagné 238 000 euros de DSU, ou encore celle de Borgo, en Corse, qui a perdu 293 000 euros de DSR et gagné 346 000 euros de DSU.

La principale entreprise du secteur, laquelle compte 250 salariés, a été placée en redressement judiciaire. Certes, la crise économique peut constituer une explication, mais il semble également que les opérateurs privés subissent les effets d'une distorsion de concurrence avec les activités de l'Institut

En juin 2017, l'Autorité de la concurrence a reconnu un risque de « subventions croisées pouvant aboutir à des prix prédateurs ou produire des effets d'éviction ». Cette instance a donc demandé à l'INRAP une séparation comptable entre ses missions de service public et ses activités commerciales. Cet engagement a-t-il été respecté depuis lors ? En outre, sachant que la loi du 17 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a régulé ce secteur, qui dépend des décisions publiques, il semble urgent de lancer une mission de l'Inspection générale des finances.

l'activité des entreprises du secteur de l'archéologie préventive s'est contractée entre 2013 et 2016, en raison d'une baisse significative des opérations à réaliser. Cette situation a conduit plusieurs acteurs à se retirer, et la principale entreprise du secteur est aujourd'hui placée en redressement judiciaire. Je peux vous assurer que les services de l'État suivent avec attention la situation de l'ensemble de ces acteurs et mettent en oeuvre les moyens dont ils disposent pour les accompagner dans ce contexte économique difficile. L'Autorité de la concurrence a été saisie en 2015 par des opérateurs privés se plaignant de pratiques de l'INRAP pouvant créer des distorsions de concurrence. Dans le cadre de cette procédure, l'INRAP s'est notamment engagé à mettre en place, au plus tard le 1 janvier 2018, une comptabilité analytique permettant d'assurer une stricte séparation comptable entre, d'une part, ses activités relevant de sa mission de service public et, de l'autre, ses activités lucratives, donc ouvertes à la concurrence. Dans sa décision du 1 juin 2017, l'Autorité de la concurrence a mis un terme à la procédure engagée contre l'INRAP. Elle a estimé que les engagements proposés répondaient aux préoccupations de concurrence exprimées et présentaient un caractère substantiel, crédible et vérifiable. Conformément à ces engagements, l'INRAP a mis en oeuvre depuis le 1 janvier 2018 un nouveau modèle de comptabilité analytique, qui a été présenté et validé lors du conseil d'administration de l'établissement du 28 mars dernier. Il relève de la seule compétence de l'Autorité de la concurrence de vérifier que la comptabilité analytique mise en place par l'INRAP correspond bien aux engagements rendus obligatoires par l'Autorité. À cette fin, l'INRAP doit transmettre à l'Autorité de la concurrence une restitution annuelle comprenant un état synthétique de la comptabilité analytique auditée, ainsi que l'attestation de conformité du système de comptabilité analytique établie par l'auditeur missionné.

De même, par sa décision du 1 juin 2017, l'Autorité de la concurrence a permis de faire l'état de la situation de la concurrence dans ce secteur. Sur le fondement de ces constats, le Gouvernement a récemment pris l'initiative de plusieurs mesures visant à prévenir toute distorsion de concurrence entre les acteurs de l'archéologie préventive, notamment en garantissant l'égal accès de tous aux documents nécessaires

Ces modalités ont été fixées par le décret du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une oeuvre de l'esprit dans un cadre lucratif, lui-même précisé par un arrêté du 25 janvier 2018.

En pratique, même s'il est nécessaire de protéger le statut des amateurs participant à un spectacle lucratif, il est clair que cette réglementation peut aboutir à l'abandon de toutes les manifestations proposant une reconstitution historique ou une mise en valeur du patrimoine.

Jusqu'à la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la pratique artistique amateur n'était pas encadrée juridiquement. Ainsi, la participation d'amateurs à des spectacles courait le risque d'être assimilée à du travail dissimulé du seul fait qu'elle avait impliqué le recours à une billetterie payante, justifié l'utilisation d'équipements professionnels

d'abord créé une dérogation à la présomption de salariat afin de sécuriser le recours à des amateurs non rémunérés lorsqu'ils interviennent dans unspectacle lucratif s'inscrivant dans le cadre d'actions d'accompagnement de la pratique artistique amateur ou d'actions pédagogiques culturelles. Le décret du 10 mai 2017 a ensuite précisé le périmètre du recours aux amateurs dans un cadre lucratif, prévoyant en particulier les plafonds de représentations que vous avez rappelés. Enfin, l'arrêté du 25 janvier 2018 a finalisé le dispositif en déterminant le contenu de la convention passée avec une collectivité par les structures mobilisant des amateurs dans un spectacle professionnel et les modalités de la télédéclaration des spectacles. Ces dispositions réglementaires encadrent donc la possibilité donnée par la loi à une entreprise de spectacle de faire appel à des amateurs sans avoir à les rémunérer

patrimoine protège ainsi la pratique amateur individuelle ou en groupement constitué intervenant dans un cadre non lucratif en lui ouvrant l'accès à la publicité, à la billetterie et aux moyens techniques professionnels.

En effet, à l'occasion du Salon des fromagers qui se tenait parallèlement au Salon international de l'agriculture, j'ai été interpellé par des représentants de la profession, dont le président de la Fédération française des fromagers, qui m'ont fait part de leur inquiétude concernant l'organisation des concours « Meilleurs ouvriers de France Une nouvelle organisation est actuellement mise en place pour ces concours. En effet, un partenaire privé- en l'occurrence, une maison d'édition -prend désormais une place importante dans l'organisation des concours ainsi que dans leur financement. leur financement. Les critères de sélection et de notation ont ainsi été modifiés. Ces concours, organisés sous l'égide du ministère de l'éducation nationale, ont pour objet la reconnaissance et la valorisation de l'excellence professionnelle. le rôle prépondérant joué par un partenaire privé dans leur organisation est difficilement compréhensible pour les professionnels du secteur, qui craignent que l'indépendance et la dimension académique de ces concours ne soient remises en question.

l'excellence en toute indépendance et en toute objectivité ? Par ailleurs, pouvez-vous m'indiquer les différents acteurs du financement de ces concours et le rôle que vous entendez laisser jouer aux nouveaux partenaires privés ? La parole

L'organisation du concours pour l'obtention du diplôme d'État « Un des meilleurs ouvriers de France » repose sur un modèle original- vous l'avez rappelé -de coopération entre partenaires publics et privés, qui réunit le ministère de l'éducation nationale et ses partenaires ministériels,

Il est financé par des subventions publiques, le ministère de l'éducation nationale étant le plus gros contributeur. Il est, dans le cadre actuel, éligible à la taxe d'apprentissage. Il peut également recevoir des dons, et perçoit des droits d'inscription des candidats. Afin de pallier une fragilité financière récurrente, le comité d'organisation a passé une convention avec le groupe Uni-éditions, société filiale du Crédit Agricole. Ce partenariat financier ne présente aucun risque d'ingérence, dans la mesure où les métiers de la banque sont totalement absents des métiers ouverts au concours.

Dans le cadre de la réglementation fixée par le ministère de l'éducation nationale, le comité a ainsi rénové ses statuts et engagé une politique de transparence sur les conditions d'organisation des épreuves relevant de sa propre responsabilité. Le COET a aussi chargé l'inspecteur général, président du jury général, de revoir l'ensemble des sujets, des référentiels et des critères d'évaluation des épreuves. L'intervention des professionnels et de leurs fédérations est essentielle pour définir les exigences professionnelles attendues et, de la sorte, le niveau et la qualité du concours.

Le comité d'organisation, en accord avec sa tutelle ministérielle, a souhaité reprendre avec les fédérations professionnelles une coopération plus rationnelle dans le cadre organisationnel et juridique imparti. Une telle coopération permet d'assurer l'équilibre entre, d'une part, le respect des règles applicables aux candidats aux diplômes de l'éducation nationale la recherche permanente d'une définition de l'excellence professionnelle dans plus de deux cents métiers. Monsieur le sénateur, j'espère avoir répondu à vos inquiétudes, notamment quant à l'absence d'interférence des acteurs privés dans le processus d'évaluation.

écologique et solidaire. Madame la secrétaire d'État, dans le cadre de la réforme de l'autorité environnementale, le préfet de région était désigné comme autorité compétente de l'État en matière d'environnement.

Une instruction ministérielle non parue au préconise que les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement fassent prononcer les avis nécessaires par la mission régionale d'autorité environnementale, en lieu et place du préfet de région, sans toutefois qu'un texte législatif ou réglementaire le permette. À ce jour, nous sommes toujours dans l'attente d'un décret désignant la nouvelle autorité environnementale.

l'évaluation environnementale permet à l'autorité compétente en la matière d'autoriser ou non un projet. Cette décision est éclairée par les conséquences envisagées dudit projet sur la santé humaine et sur l'environnement. Le droit français prévoit qu'une autorité environnementale rend un avis sur le dossier en amont de l'ouverture de l'enquête publique, en indiquant comment le demandeur intègre les enjeux environnementaux dans la conception de son projet. Le 6 décembre 2017, le Conseil d'État a annulé les dispositions du code de l'environnement qui instituaient le préfet de région comme autorité compétente pour rendre l'avis d'autorité environnementale et autoriser ou non un projet.

En parallèle, le Gouvernement travaille activement à l'élaboration d'un nouveau décret. Plusieurs pistes ont été explorées pour mettre en place un dispositif à la fois conforme au droit européen et opérationnel sur le terrain. Le Gouvernement envisage une parution du décret dans le courant de l'été.

écologique et solidaire. Ma question porte sur le coût de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides.

puis, dans un second temps, les produits contenant ces substances actives ayant vocation à être commercialisés en France doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. L'instruction de cette demande par l'ANSES a un coût, qui est à la charge des entreprises souhaitant commercialiser des produits biocides. Son montant est fixé, par arrêté, de manière forfaitaire et par produit contenant des substances actives. ce mode de calcul forfaitaire et par produit, indépendant de la quantité produite. En effet, le coût d'instruction pour la commercialisation d'un produit est le même que ce dernier soit commercialisé par un grand groupe et à l'échelle nationale, ou bien par une petite entreprise dont le réseau de diffusion n'est que régional, voire départemental. En vertu du principe du pollueur-payeur, il semblerait plus juste qu'une entreprise produisant des centaines de milliers de tonnes

Ce texte a été élaboré en concertation avec les organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine des produits biocides. Il n'a pas été jugé pertinent de moduler le montant de la redevance en fonction de la taille de l'entreprise, car les frais engagés par les pétitionnaires servent à couvrir les coûts de l'instruction

qui n'existent pas dans d'autres pays européens ; je pense par exemple au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt innovation. Ce dernier, consacré spécifiquement aux TPE et PME, leur permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 20

Je vous remercie

écologique et solidaire. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur la diminution des aides publiques destinées à l'électrification rurale et, plus précisément, sur la situation du syndicat départemental d'énergie du Calvados, le SDEC Énergie.

La priorité du SDEC Énergie est naturellement le renouvellement des installations électriques obsolètes et le renforcement du réseau. Or, avec une dotation du FACÉ amputée de 20 %, notre syndicat départemental ne pourra plus continuer à investir et, à court terme, la qualité du réseau d'électricité en secteur rural en sera affectée. Cette situation est d'autant plus mal vécue que l'inventaire de l'état du réseau apparaît tronqué. En effet, depuis plusieurs années, le SDEC Énergie réalise à sa charge des campagnes de mesure de tension qui, sur la base de plusieurs centaines d'enregistrements, démontrent une différence notable- de plus de 20 %, tout de même -entre la mesure réalisée chez l'habitant et l'étude statistique GDO d'Enedis.

attention sur la problématique des écarts de mesure de tension que je viens d'évoquer, et souhaite également connaître votre position sur cette question. Enfin, plus globalement, pourriez-vous préciser les intentions du Gouvernement quant à l'avenir du FACÉ ? Une augmentation de cette aide publique à l'électrification rurale est-elle envisagée pour 2019 ? La parole

comme vous le soulignez, le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, le FACÉ, doté de 360 millions d'euros en 2018, permet de réaliser les investissements nécessaires pour la qualité du réseau de distribution d'électricité en milieu rural. Cet outil essentiel

un inventaire de l'état de nos réseaux électriques qui nous a permis de démontrer l'efficacité du FACÉ et l'amélioration continue de la qualité de la redistribution d'électricité en milieu rural. Ainsi, pour l'année 2018, la dotation du syndicat départemental d'énergie du Calvados s'élève à plus de 5 Elle était de 6,4 millions d'euros en 2017. Cette diminution est le produit de deux effets, l'un contextuel et l'autre factuel. Premièrement, lapolitique d'électrification rurale participe, comme l'ensemble des politiques publiques, à l'effort de redressement des finances publiques. Dans ce cadre, le montant total du FACÉ, voté dans la loi de finances pour 2018, est en baisse de 5 %, passant à 360 millions d'euros. Deuxièmement, en ce qui concerne les zones rurales du Calvados, le dernier inventaire a établi l'évolution favorable de la qualité du réseau électrique basse tension. À l'inverse, les

ont par ailleurs été approuvés à l'unanimité par le comité compétent. La diminution de 20 % des dotations octroyées au Calvados résulte donc d'un arbitrage que nous jugeons juste, équitable et transparent. La

tronquée de la réalité du réseau et de la qualité de l'électricité distribuée dans le département. Sachez, madame la secrétaire d'État, que je me tiens à votre disposition, de même que les responsables du SDEC Énergie, pour travailler sur ces questions. L'électrification en milieu rural, notamment dans un département comme le mien, est un enjeu

chargée des transports. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur l'aménagement de l'autoroute A8, qui passe à proximité de la commune de Biot, dans les Alpes-Maritimes,

les buses de l'autoroute A8, gérée sur le réseau Escota par Vinci Autoroutes, se sont bouchées, empêchant l'eau de s'écouler normalement. L'eau a alors stagné à une hauteur de plus de 1,50 mètre, pendant plus d'une heure, dans des zones d'habitation de la commune de Biot. de la commune de Biot. En mars 2018, lors d'une intempérie sans conséquence, puisque sa puissance n'a été décelée ni par la préfecture, ni par Météo France, ni par les logiciels municipaux, le même schéma s'est reproduit.

Pris au piège par l'eau dans la zone de rétention, les habitants n'auraient eu aucun moyen de fuir, sans parler des dommages matériels subis que nous aurions pu répertorier une fois de plus, notamment sur les habitations. Après les intempéries de 2015, la maire de Biot, Mme Guilaine Debras, avait alerté, sans succès, le précédent gouvernement, ainsi que le concessionnaire autoroutier, Vinci, afin de discuter des aménagements qu'il faudrait apporter à cette autoroute, qui forme un véritable barrage à l'écoulement de l'eau en cas de fortes pluies. Madame la secrétaire d'État, si Vinci est gestionnaire d'Escota, l'autoroute reste bien la propriété de l'État. Comptez-vous donc intervenir auprès du concessionnaire afin de réduire le risque d'inondation en ordonnant les travaux d'aménagement nécessaires à la sécurité des habitants et à la pérennité des infrastructures ?

nous partageons vos préoccupations. Sur la base des discussions engagées autour du bassin de la Brague entre les collectivités territoriales, les services de l'État et la société Escota, concessionnaire de l'autoroute A8, une étude hydraulique a été commandée en 2015 par la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Cette étude a été transmise aux services du ministère des transports, où elle est en cours d'analyse,

ni de l'accentuation des phénomènes d'engorgement. Ils ont en conséquence aggravé le phénomène d'écoulement des eaux au droit des ouvrages de l'autoroute A8. La situation n'est donc pas satisfaisante ; nous partageons ce constat avec vous. Soucieuse Soucieuse de l'amélioration de la situation et de la garantie apportée à la sécurité des personnes, Élisabeth Borne a demandé elle-même à ses services de traiter ce dossier avec vigilance. Le programme d'aménagement devra être examiné au regard des conditions permettant de limiter les incidences sur les populations et territoires en aval de l'autoroute.

dans un cursus universitaire, par le biais de la capacité en droit. Or ces étudiants ne sont pas traités de manière égalitaire, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une bourse, ni en première ni en seconde années.

cette raison, la capacité en droit ne fait pas partie des formations ouvrant droit au bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Pour autant, le public de cette formation n'est pas dénué de droits, et le Gouvernement travaille à les renforcer. En matière de protection sociale, les étudiants inscrits en capacité en droit ne seront plus assujettis au régime de la protection sociale des étudiants, qui est voué à disparaître conformément aux dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. des étudiants. Ils seront désormais affiliés, en tant qu'assurés autonomes, à leur régime de protection sociale, généralement celui de leurs parents, c'est-à-dire le régime général de la sécurité sociale. La cotisation annuelle de 217 euros sera supprimée pour tous les nouveaux étudiants dès la rentrée 2018 ; elle le sera pour l'ensemble des étudiants en 2019. Les étudiants inscrits en capacité en droit bénéficieront de cette mesure générale, qui se traduira par un gain net de pouvoir d'achat dès la rentrée prochaine.

Le gel des salaires depuis 2010 entraîne une précarisation accrue de ces agents, dont une grande partie perçoit la prime d'activité. Les départs en retraite non remplacés et la multiplication des contrats précaires, avec recours aux heures supplémentaires comme variable d'ajustement, creusent le manque d'effectifs et accentuent la détérioration des conditions de travail. Les agents font aussi face à un management dont la boussole est la rentabilité. Des missions sont mutualisées et externalisées, au détriment de la qualité du traitement des dossiers et du service rendu aux usagers. Ainsi, la paie des agents de Seine-Saint-Denis est traitée à Paris, tandis que des traitements de données sont confiés à des entreprises privées. Malgré l'augmentation des charges de travail et la complexité accrue de la législation, les agents n'ont aucune reconnaissance de leur métier. Par ailleurs, les fermetures de locaux contraignent les agents, mais aussi les familles, à se déplacer régulièrement, aux dépens d'un service de proximité. Les conventions d'objectifs et de gestion se succèdent, toujours plus drastiques. Les organismes sont de plus en plus sous tension dans l'ensemble des branches, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où, de ce fait, de nombreuses familles ne peuvent être accompagnées.

a moins de tout, le Gouvernement va-t-il prendre les mesures qui s'imposent pour que les caisses d'allocations familiales puissent accomplir au mieux leurs missions ? La parole

en lieu et place de ma collègue ministre des solidarités et de la santé, qui ne peut être ici ce matin. La caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, au regard de l'augmentation du nombre de bénéficiaires, est victime d'un allongement des délais de traitement des dossiers.

Des milliers de stades, qui appartiennent le plus souvent aux communes, sont couverts d'une très grande quantité de granulats issus du recyclage de pneus broyés. Ces substances seraient, selon plusieurs études récentes, fortement nocives à la fois pour la santé, de la présence de composés hautement cancérogènes, et pour l'environnement. Des solutions existent, telles que l'aspiration des billes et le remplacement par des matériaux naturels, ou encore l'encapsulement par résine, mais elles présentent un coût élevé. En outre, de nombreux terrains sont en commande ou en cours d'installation, et le simple report envisagé par certains élus entraîne lui aussi des frais colossaux. Interpellée par plusieurs parlementaires, Mme la ministre des sports a répondu en des termes ambigus, pointant à la fois des études rassurantes et des incertitudes, avec pour conséquence la saisine par six ministères de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'ANSES devrait rendre très prochainement Selon les données invoquées, qui ont d'ailleurs été très largement contredites, les risques pour la santé seraient négligeables, du fait d'un seuil de toxicité en accord avec les normes européennes.

du principe de précaution, il ne faut pas, en présence d'un risque de dommages graves et irréversibles, que l'absence de certitude scientifique absolue serve de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives. C'est pourquoi je demande au Gouvernement de mettre en place un fonds d'urgence à destination des collectivités territoriales, afin de les aider à engager des travaux de mise en sécurité de leurs équipements, à reporter leurs marchés publics dans l'attente des conclusions de l'ANSES

Ces terrains synthétiques soulèvent des interrogations quant à leurs effets sur la santé et l'environnement en raison de substances dangereuses potentiellement présentes dans des granulés, en particulier dans le cadre de leur utilisation comme terrain de sport ou aire de jeux pour enfants. L'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, a conclu à un faible niveau de préoccupation, au vu des concentrations d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il faut toutefois remarquer que les limites de concentration prévues par le règlement REACH ne sont pas spécifiques à un usage pour des terrains synthétiques, ce qui soulève, il est vrai, des incertitudes. Face aux préoccupations des pratiquants et des communes, principaux propriétaires de terrains de grands jeux dans notre pays, les ministères de la transition écologique et solidaire, des solidarités et de la santé, de l'économie et des finances, du travail, de l'agriculture et de l'alimentation, et des sports, ont saisi l'ANSES le 21 février dernier. Dans un premier temps, l'ANSES fera part de son analyse sur les données et études disponibles, ainsi que sur les préoccupations qui pourraient en résulter. La publication de ce premier travail est attendue pour la fin du Dans un second temps, l'Agence devra compléter son analyse en identifiant et en hiérarchisant les besoins de connaissances supplémentaires qui pourraient justifier une évaluation des risques pour la santé et l'environnement à plus long terme. Nous ne manquerons pas, madame la sénatrice, de vous communiquer les résultats de ces travaux.

je me permets d'insister, parce que je ne voudrais pas que, dans quelques années, on nous accuse, on vous accuse, d'avoir laissé passer un risque sanitaire et environnemental majeur- cancers, asthme et autres pathologies respiratoires, mais aussi diffusion dans l'atmosphère -dont nous découvrirons sûrement rapidement les effets.

dans sa commune, selon son propre intérêt sur la question, mais aussi selon ses moyens financiers et les remontées des usagers- parents, professeurs, ou associations, de futsal, par exemple. Enverrez-vous des instructions claires aux communes,

fait du manque de médecins généralistes et des nombreux départs à la retraite, de plus en plus de patients se retrouvent aujourd'hui sans médecin traitant. Ils vivent cette situation subie avec d'autant plus d'inquiétude, voire d'angoisse, qu'ils sont vulnérables, malades, âgés ou isolés.

L'accès aux soins repose, non pas sur l'installation d'un médecin, mais sur l'organisation coordonnée de tous les professionnels de santé d'un territoire donné. C'est pourquoi nous travaillons actuellement sur la stratégie du système de santé. Le plan comme la stratégie ont pour objectif d'augmenter le temps soignant des professionnels de santé ; ils généralisent la téléconsultation et la téléexpertise. Mme Buzyn l'a toujours dit : ce plan sera amené à évoluer en fonction des besoins. Voilà pourquoi, à la suite des derniers chiffres de la souhaite le compléter par de nouvelles mesures. Votre proposition est une demande forte et légitime des patients, qu'il faut étudier. Pour remédier aux difficultés auxquelles font face nos concitoyens en matière d'accès aux soins, il n'y a pas de réponse miracle, mais un panel de solutions. Ces solutions, c'est ensemble que nous devons les trouver ! La parole

C'est ainsi que, depuis 2008, les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l'exception de la primo-vaccination.

de vaccination, ce qui limite la couverture vaccinale. De nombreux rapports ont préconisé, pour assurer une couverture vaccinale large, une simplification de la vaccination en ville, notamment la possibilité pour les professionnels de santé autres que les médecins

et efficace. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle permet d'éviter deux à trois millions de décès chaque année dans le monde pour les seules maladies de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche et de la rougeole. Acteurs majeurs de la prévention et du soin, les infirmiers peuvent, sur prescription médicale, vacciner la population générale pour tous les vaccins. Depuis 2008, ils peuvent aussi vacciner sans prescription médicale- à l'exception des primovaccinés et des femmes enceintes -les personnes cibles de la vaccination antigrippale, à savoir les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et les patients porteurs de pathologies chroniques comme les infections cardio-pulmonaires, le diabète ou l'obésité. cette possibilité offerte aux infirmiers. Compte tenu des résultats encourageants enregistrés, Agnès Buzyn a souhaité conduire une réflexion sur l'élargissement des compétences des infirmiers en matière de vaccination, afin de simplifier et d'améliorer le parcours vaccinal d'un plus grand nombre de personnes.

Elle continue notamment à prendre insuffisamment en compte toutes les prévisions démographiques faisant systématiquement état d'un allongement de la durée de vie dans l'Hexagone. Aussi, et en dépit d'avancées certaines portées par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la situation est aujourd'hui particulièrement préoccupante. Le nombre trop réduit d'établissements spécialisés en gériatrie

de pouvoir mener à bien leur mission. Il n'en demeure pas moins que ces établissements sont littéralement pris d'assaut. C'est notamment le cas des établissements implantés dans le Nord lorrain, dont certains disposent d'une unité Alzheimer. Malheureusement, leur capacité d'accueil est limitée : toutes leurs chambres sont aujourd'hui occupées. Ouvrir un nouvel établissement serait naturellement la solution idéale. Or, du point de vue financier, la création d'un EHPAD représente un investissement important, même dans le cadre d'un partenariat public-privé. d'un nouvel établissement est à l'étude- et toujours seulement à l'étude -à Ars-sur-Moselle, commune qui attend depuis plusieurs années maintenant la construction d'un EHPAD. Cette situation n'étant pas spécifique à la Moselle,

réponds en lieu et place de Mme la ministre des solidarités et de la santé. Nous sommes face à un véritable enjeu de société. Vous avez raison, nous devons changer en profondeur le modèle des EHPAD en tirant le meilleur parti de ce qui se fait déjà dans les territoires. L'augmentation du nombre de places d'hébergement temporaire est également nécessaire, et nous devons mieux les valoriser financièrement. L'une des priorités de Mme Buzyn sera de valoriser les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées, notamment en orientant les nouveaux contrats parcours emploi compétences vers les EHPAD.

présentent un état de santé de plus en plus compliqué à soigner. Or les dotations en soins ne suivent pas, ce qui engendre un manque de personnel et, d'une certaine manière, une forme de maltraitance.

La séance est reprise.

ministre de la justice. Madame la ministre, en tant qu'élue des Français établis hors de France, je suis très souvent sollicitée pour résoudre des difficultés rencontrées dans le cadre de démarches d'obtention d'un certificat de nationalité française.

En 2014 déjà, des mesures d'urgence avaient été mises en place, et des renforts temporaires accordés. Malgré cela, le retard accumulé n'a manifestement pas été absorbé, puisqu'il faut compter en moyenne trois ans de procédure, au lieu de deux ans. Cette situation n'est pas acceptable : imaginez la détresse de la personne que l'on informe du temps moyen qu'il faut attendre pour faire reconnaître la nationalité française de son enfant et pouvoir le faire venir en France

Ma question est la suivante : des mesures d'urgence comme des mesures pérennes vont-elles être mises en place afin de garantir un réel service public de la justice ? Si oui, lesquelles et, surtout, quand ?

000 demandes de délivrance de certificats de nationalité sont enregistrées chaque année dans les tribunaux d'instance. Près d'un tiers des certificats sont délivrés à Paris. Les délais de délivrance que vous avez relevés, et qui sont effectivement très longs, ont deux explications principales

un droit très ancien peut trouver à s'appliquer, auquel cas il faut parfois remonter toute une chaîne d'ascendants pour trouver l'ascendant français transmettant sa nationalité et, donc, le droit qui s'applique. outre, pour les personnes originaires de territoires devenus indépendants, il faut vérifier les conditions de conservation et de perte de la nationalité française qui ont été fixées par les traités signés lors des indépendances, ce qui peut parfois prendre un certain temps. Par ailleurs, au sens de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité repose sur celui qui s'en prévaut. Il appartient donc au demandeur de réunir et de déposer les pièces qui sont liées à sa demande. Chaque situation étant unique, je le répète, le requérant se voit par conséquent chargé

que certaines erreurs relevées peuvent également faire l'objet de jugements de rectification des actes demandés. Cependant, les preuves doivent être délivrées par l'autorité étrangère compétente et être complétées par la transmission d'un nouvel acte qui porte la mention de la rectification dudit

Outre la complexité des demandes et leur nombre, le délai de délivrance résulte également de difficultés qui peuvent être liées à un certain manque d'effectifs dans les juridictions. Cette situation va s'améliorer

Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions. Pour avoir visité le service de la nationalité, rue du Château-des-Rentiers, à Paris, et pour avoir parlé à son directeur, je suis bien consciente de la complexité des procédures.

Madame le ministre, les différentes modifications législatives intervenues l'an dernier en matière de gestion et de contrôle des partis politiques

Malheureusement, il est difficile d'obtenir des réponses précises, aussi bien de la part de l'administration que de la part de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

constitués », entre autres, « des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ». La CNCCFP précise que, pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, elle a recours à la technique du faisceau d'indices développée par le juge financier et le juge administratif à l'encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives. la CNCCFP examine si le parti politique est à l'initiative de la création de l'entité, en contrôle l'organisation et le fonctionnement, et lui procure l'essentiel de ses ressources. Dans l'affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l'entité doivent être consolidés dans les comptes d'ensemble du parti. Dans ce contexte, et pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, l'aide financière attribuée par un parti politique à un tiers ayant ou non un objet politique, relevant ou non de la loi du 11 mars 1988, sera analysée analysée pour les comptes de l'exercice 2017 au regard de ces différents critères, et non au seul regard de la dépendance financière de l'un envers l'autre. Enfin, en application du décret du 28 décembre 2017 pris pour l'application de la loi pour la confiance dans la vie politique, le périmètre des comptes d'ensemble des partis pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017 devra inclure les comptes des organisations territoriales affiliées au parti, avec son accord ou à sa demande, ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne. À cet égard, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi précitée, l'Autorité des normes comptables doit établir un projet de règlement dont la version définitive devra être homologuée par le ministre de l'économie et des finances avant la fin de l'année 2018.

occasion prendre un grand nombre de décisions en moins de vingt-quatre heures. C'est pourquoi la transparence quant au coût

qui nous concerne évidemment tous. Les familles venant de perdre un être cher sont malheureusement amenées à prendre des décisions importantes, dans un temps extrêmement contraint et à un moment particulièrement difficile. Votre proposition de loi, loi, devenue la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, a incontestablement constitué une avancée très importante. Elle a notamment instauré, vous l'indiquiez, un modèle de devis pour les prestations funéraires. L'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, qui a été modifié par l'arrêté du 3 août 2011, est ensuite venu définir une terminologie commune, permettant de faciliter la comparaison des tarifs pratiqués par les différentes entreprises de pompes funèbres. Ce modèle de devis est en vigueur depuis le 1 janvier 2011 et il a permis aux familles d'organiser les obsèques de leurs proches dans une plus grande transparence des prix et des pratiques commerciales. également mentionné une enquête publiée par l'association Familles rurales le 1 novembre 2017, selon laquelle 4 entreprises habilitées sur 10, seulement, respectent cette obligation. Comme vous, je ne peux que déplorer ce résultat. La situation décrite par cette enquête ne peut pas perdurer. L'application de la loi doit devenir effective sur l'ensemble du territoire. Dans ces conditions, le Gouvernement va travailler à renforcer le dispositif de contrôle du respect de cette obligation, ainsi que le dispositif de sanctions en cas de manquement. Ces devis étant consultés selon les modalités définies dans chaque commune par le maire, j'ai également souhaité que les représentants des collectivités siégeant au sein du Conseil national des opérations funéraires soient à nouveau sensibilisés sur l'importance de l'application de ces dispositions et qu'ils veillent à faciliter cette mise en oeuvre. Ce sera fait

il serait naturel que les préfets- et à cet égard, le ministère de l'intérieur peut donner des instructions -retirent ou suspendent l'habilitation. Je vous assure qu'une telle mesure, très simple, aurait des effets très concrets.

de l'intérieur. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur les conséquences de la contractualisation entre les collectivités territoriales et l'État. La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 dispose que « les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique ». Sur le fondement de ce texte, le Gouvernement propose aux collectivités une contractualisation visant à encadrer leurs dépenses de fonctionnement, avec une marge de progression très serrée. La loi précise en effet que l'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 %, appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant, sur les cinq années concernées. Pour le conseil départemental de la Haute-Savoie, ce cadrage laisse une marge de 7 millions d'euros de dépenses de fonctionnement pour chaque année. Or notre département connaît, depuis deux décennies, une progression démographique particulièrement forte, de l'ordre de 1,2 %. Plus précisément, ce sont 10 000 habitants

De plus, je tiens à souligner un point important : la seule prise en charge des mineurs non accompagnés, les MNA, absorbe annuellement une enveloppe de 4 millions d'euros. Ainsi, l'objectif d'encadrement des dépenses de fonctionnement proposé par le Gouvernement apparaît strictement impossible à atteindre, et ce alors même que le département se montre, depuis plus d'une décennie, exemplaire dans la gestion de ses finances. À titre d'exemple, il respecte un ratio entre le nombre de fonctionnaires territoriaux et et la population très inférieur à la moyenne nationale et s'attache à parvenir à un taux d'endettement parmi les plus faibles de France. En matière de maîtrise des dépenses, un effort considérable a été

En conclusion, alors que le département de la Haute-Savoie atteint pleinement les objectifs de désendettement affichés comme prioritaires par le Gouvernement, il se trouve durement pénalisé par l'exigence qui est lui est faite de financer un volet de la politique migratoire. Il est nécessaire, à mon sens, de prendre en compte de telles situations et de prévoir des dispositions dérogatoires pour les collectivités, dont le nombre est d'ailleurs limité, qui y sont confrontées. Je vous demande donc, madame la ministre, de bien vouloir m'indiquer les mesures que le Gouvernement

Monsieur le sénateur Carle, vous appelez mon attention sur le dispositif des contrats de maîtrise de la dépense entre l'État et les collectivités, représentant les deux tiers de la dépense publique locale. Ce dispositif constitue un axe majeur de la nouvelle relation de confiance que le Gouvernement souhaite établir avec les collectivités, notamment avec les départements. C'est bien dans cet état d'esprit qu'il a été conçu, aux termes d'échanges nourris avec les représentations d'élus. Ces discussions ont permis d'aboutir à un mécanisme prenant en compte les spécificités de chacune des collectivités concernées. concernées. À ce titre, personne ne peut nier que, comme vous le faites remarquer, une augmentation de la population engendre des charges supplémentaires. L'article 29 de la loi de programmation mentionnée par vos soins permet de tenir compte de ce phénomène. Il ouvre en effet la possibilité d'une modulation à la hausse du taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement figurant dans le contrat d'au plus 0,15 point pour les collectivités connaissant une progression démographique marquée. Le département dont vous êtes l'élu est bien éligible à cette modulation, sa population ayant augmenté, en moyenne, de près de 1,5 % entre 2013 et 2018. Vous mentionnez par ailleurs la problématique des MNA pris en charge par les conseils départementaux au titre de l'aide sociale à l'enfance. Vous le savez, le Gouvernement est pleinement conscient de l'acuité de ce phénomène et des dépenses qu'il peut entraîner. Des négociations ont eu lieu avec l'Assemblée des départements de France et une solution, je crois, est en train d'être trouvée, portant sur la reprise par l'État du dispositif d'évaluation et sur une participation au niveau du dispositif de prise en charge post-évaluation. Nous sommes évidemment sensibles aux efforts que les départements doivent continuer d'accomplir dans ce domaine. C'est pour cette raison qu'une négociation a été engagée avec les représentants des départements, en vue d'un accord global sur le financement des allocations individuelles de solidarité, les mesures financières supplémentaires pour les MNA et sur l'application qui peut en être faite en cas d'augmentation de ces dépenses dans les contrats. Je souhaite enfin vous rappeler que les contrats ne se résument pas à la fixation d'un objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement. Les échanges avec le préfet sur l'amélioration du besoin de financement financement permettront de mettre en lumière les engagements de votre département en matière de bonne gestion de ses finances, de même que des éléments d'explication d'ordre qualitatif- les élus locaux peuvent, s'ils le souhaitent, en faire figurer dans ces mêmes contrats.

de l'Isère Olivier Véran, les communes dont les habitants ont accouché ou sont décédés dans un établissement situé hors du territoire communal contribuent aux charges de tenue de l'état civil de la commune siège dudit établissement, selon trois critères de seuil. Sont pris en compte dans ce cadre la taille de la commune accueillant l'établissement, le rapport entre le nombre de naissances dans l'établissement et la population de la commune qui l'accueille et, enfin, le nombre de décès ou de naissances imputables, si je puis dire, aux habitants des communes appelées à contribuer aux charges.

contribution. La commune d'accueil du centre hospitalier supporte ainsi, de fait, une charge très largement supérieure à celle qui devrait être la sienne, eu égard au nombre de ses propres habitants nés ou décédés dans l'établissement de santé. À titre d'exemple, dans mon département, la commune de La Tronche- hospitalier universitaire de Grenoble. En 2016, près de 3 000 enfants y sont nés et 2 000 personnes y sont décédées. La mairie traite plus de 54 000 actes par an, maintient un service composé de 9 agents, pour une charge budgétaire représentant près de 350 000 euros. Si La Tronche ne devait supporter que les actes induits par les naissances et décès de ses propres habitants, sa charge budgétaire 6 588 euros ! La commune n'est pas seule dans ce cas. Rien qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, mes collègues de la Loire, avec Saint-Priest-en-Jarez, du Rhône, avec Pierre-Bénite, ou encore de Haute-Savoie, avec Metz-Tessy, pourraient sans doute en témoigner. Il apparaît dès lors qu'une fixation de ce seuil à 0,1 %, plutôt qu'à 1 %, permettrait une répartition beaucoup plus équitable. Madame la garde des sceaux, de quelle manière le Gouvernement pourrait-il envisager une modification de cette répartition des charges,

Cette contribution a été créée par la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Elle s'appliquait initialement selon les trois critères de seuil suivants : la différence entre le nombre de naissances comptabilisées au sein de l'établissement et la et la population d'implantation devait dépasser 40 % ; la commune dans laquelle se situait l'établissement devait compter moins de 3 500 habitants ; la contribution financière s'appliquait seulement aux communes dont les habitants représentaient au moins 10 % des naissances ou des décès constatés dans l'établissement. L'intention du législateur était donc de répondre aux situations exceptionnelles de petites communes situées à proximité de grandes villes et accueillant de grands hôpitaux. La loi NOTRe a étendu ce dispositif, pour prendre en compte la hausse des charges d'état civil d'un plus grand nombre de petites communes en difficultés financières. Le plafond des communes éligibles au dispositif a été rehaussé pour englober toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Le seuil d'éligibilité entre les naissances constatées dans un établissement et la population d'implantation a été abaissé à 30 %. Enfin, la contribution financière des communes extérieures a sensiblement augmenté, puisqu'elle s'applique à toutes les communes ayant plus de 1 % de naissances ou de décès dans un établissement.

des dernières années, les missions dévolues par les municipalités à leur police municipale ont eu tendance à s'étoffer, en raison des événements survenus en France et de la menace terroriste qui pèse sur notre pays. Les policiers municipaux ont incontestablement gagné en professionnalisme et assurent une sécurité de proximité indispensable et complémentaire à l'intervention de la police nationale. Pourtant, ils ont de grandes difficultés à assurer ces missions dans des conditions décentes, car les moyens dont ils disposent sont limités. Par exemple, lors d'un banal contrôle de vitesse, ils n'ont pas accès au fichier national des permis de conduire- le FNPC -pour s'assurer de la détention effective et de la validité du titre présenté, ni au fichier des véhicules volés- -avant de procéder à la mise en fourrière d'un véhicule, ni au système d'immatriculation des véhicules- le SIV -pour notifier l'immobilisation ou l'annulation de l'immobilisation d'un véhicule, ni au fichier des personnes recherchées- qui permettrait également de garantir des conditions d'intervention plus sûres, notamment dans cette période de menace terroriste. sont donc dans l'obligation de faire appel à leurs collègues de la police nationale ou de la gendarmerie pour pouvoir effectuer toutes les vérifications d'usage qui s'imposent, même pour un banal contrôle de vitesse. Il s'agit incontestablement d'une perte de temps et d'efficacité pour la police nationale, comme pour la police municipale, qui ne dispose pas de tous les moyens indispensables au bon accomplissement de ses missions. C'est pourquoi de nombreux élus m'ont demandé d'intervenir ce matin. Ils souhaiteraient que l'État puisse revoir sa position concernant

Une personne ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de sa fonction. Dès lors que les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints, ne disposent pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'y a pas nécessité de leur ouvrir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder. Ainsi, au regard des missions dévolues aux policiers municipaux, il n'a pas été jugé nécessaire de leur permettre un accès direct au fichier des personnes recherchées, le FPR. Je tiens à vous rappeler qu'en application des dispositions en vigueur les policiers municipaux peuvent déjà être rendus destinataires, sous certaines conditions, d'informations issues de ce fichier, notamment afin de parer à un danger pour la population. Pour des raisons similaires, un accès direct des policiers municipaux au fichier des objets et des véhicules signalés, le FOVeS, qui a remplacé le fichier des véhicules volés, Dans la pratique, les agents de police municipale peuvent avoir accès à un extrait actualisé du fichier en saisissant la plaque d'immatriculation sur leur terminal personnel, afin de savoir si un véhicule est volé ou utilise des plaques aux numéros usurpés avant mise en fourrière. outre, le Gouvernement ne peut que vous rejoindre sur la nécessité d'ouvrir aux agents de police municipaux un accès direct au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire,

parlementaire en cours sur le continuum de sécurité, portée par les députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, nous apportera un éclairage intéressant sur l'adaptation des conditions d'accès des policiers municipaux à ces fichiers.

ministre de l'intérieur. Madame la ministre, je me permets d'attirer votre attention sur la demande d'effectifs nécessaires dans les commissariats de police de Vendée. Par un courrier en date du 2 novembre 2017, dont vous avez accusé réception, je vous ai alertée sur les conditions de travail dégradées dans les commissariats de La Roche-sur-Yon et des et des Sables-d'Olonne. Le 8 février dernier, vous avez annoncé le lancement de la police de sécurité du quotidien- ou PSQ -, plan quinquennal ambitieux qui vise à construire dans notre pays une société rassemblée et apaisée. En Vendée, la mise en place de cette police de sécurité du quotidien devait conduire à l'arrivée d'effectifs supplémentaires à la gendarmerie de Fontenay-le-Comte, mais rien n'était envisagé pour les commissariats de police des Sables-d'Olonne et de La Roche-sur-Yon. Or si ces établissements ne sont pas directement concernés par le nouveau dispositif, le besoin de personnel complémentaire n'en est pas moins indispensable. La Vendée fait partie des 20 départements dans lesquels les extractions judiciaires sont toujours assurées par les

à ce jour. Mais, surtout, les effectifs de référence sont totalement obsolètes et la situation ne s'arrange pas, avec un nombre de résidents qui continue d'évoluer à la hausse. hausse. La carence en personnel se concrétise par des journées à rallonge, des décalages horaires incessants. Le taux d'effectif en arrêt de travail ou en mi-temps thérapeutique atteint 20 % ! Depuis l'annonce du 8 février, la situation a évolué et je vous remercie d'avoir répondu aux attentes du commissariat des Sables-d'Olonne. délits soient constatées, comme l'outrage sexiste du projet de loi de la secrétaire d'État Marlène Schiappa, les commissariats doivent être suffisamment dotés en personnel. Le 2 juillet prochain, la commission administrative paritaire nationale statuera sur les mutations.

en Vendée. La sécurité, vous le savez, est une priorité pour ce gouvernement et, en la matière, les attentes des Français sont grandes, qu'il s'agisse de terrorisme ou de délinquance du quotidien. C'est pourquoi, dans un contexte budgétaire contraint, le Gouvernement a fait le choix de renforcer les moyens matériels et humains des forces de l'ordre, avec, notamment, le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes au cours

couplées à une simplification significative, écrit mon collègue de l'Intérieur, de la procédure pénale à venir- j'en suis d'accord. Si les effectifs de police en Vendée ont légèrement diminué entre 2016 et 2017, le nombre de gradés et de gardiens de la paix affectés en sécurité publique- ce sont les principaux policiers mobilisés au quotidien sur la voie publique -est, lui, quasi conforme à l'effectif de référence de ce département. On dénombre 153 personnels, pour un effectif cible de 154. La circonscription de police de La Roche-sur-Yon compte, elle, 125 agents, avec un nombre de gradés et de gardiens de la paix très légèrement supérieur à l'effectif de référence, dont je sais- M. le maire me l'a dit -qu'il est contesté.

à une unité près, à son effectif de référence. J'ajoute qu'un poste d'officier de police judiciaire y a été ouvert au titre du mouvement de mutation dit « profilé » pour une prise de poste au 1 septembre 2018. Comme pour La Roche-sur-Yon, la situation des effectifs de cette circonscription sera réexaminée dans le cadre du mouvement de mutation polyvalent 2018. Vous pouvez être certaine, madame la sénatrice, qu'en Vendée comme sur l'ensemble du territoire national, tout sera fait pour doter les forces de l'ordre des moyens et des modes d'action qui leur permettront d'être très proches du terrain et d'agir efficacement. Bien sûr, l'implication des élus locaux, dont je peux porter témoignage, sera, elle aussi, l'une des clés de la réussite.

et, dans ce cadre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés que rencontrent les présidents et vice-présidents de communautés de communes, faute d'être remboursés de leurs frais de transport au sein des Les modalités de remboursement de ces frais sont actuellement régies par le code général des collectivités territoriales, le CGCT. Les conseillers d'EPCI ne sont remboursés de leurs frais de transport que s'ils ne touchent pas d'indemnité dans le cadre de leur fonction et si le déplacement a lieu en dehors de leur commune. De fait, les présidents et vice-présidents d'EPCI percevant une indemnité ne peuvent donc pas bénéficier de ces remboursements. Ces dispositions ne sont pas adaptées à la réalité de notre territoire. En effet, les EPCI ont souvent une superficie très étendue, mais comptent peu d'habitants, ce qui implique des indemnités faibles pour leurs présidents et vice-présidents. Ma communauté de communes, par exemple, a un diamètre de 100 kilomètres pour 38 000 habitants. Les président et vice-présidents touchent donc un peu plus de 1 000 euros par mois et doivent parcourir des distances considérables pour accomplir leur devoir de représentant communautaire. Leur indemnité est alors uniquement dédiée à leurs frais d'essence, ce qui est contraire à son esprit originel. Ainsi, madame la ministre, pouvez-vous envisager la mise en place d'un système de remboursement des frais de transport pour les présidents et vice-présidents de communautés de communes sur justificatifs, comme cela existe d'ores et déjà pour les conseillers régionaux ? Très bonne question ! La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

qui ne bénéficient pas d'une indemnité de fonction au titre de leur mandat intercommunal peuvent demander l'indemnisation des frais de déplacement engagés à l'occasion de certaines réunions qui ont lieu dans une commune autre que la leur. Le législateur n'a pas entendu autoriser le remboursement des frais de déplacement aux élus des communautés de communes qui bénéficient d'une indemnité de fonction. Lors de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, le Sénat avait repoussé un amendement qui tendait à leur accorder ce remboursement, après un débat qui avait été particulièrement intense. Les arguments échangés étaient alors les mêmes qu'aujourd'hui. En revanche, les élus des communautés de communes peuvent, en application de l'article L. 5211-14 du CGCT, être remboursés des frais engagés lors de l'exécution d'un mandat spécial, dans les mêmes conditions que les élus municipaux. Vous avez raison de souligner la difficulté engendrée par ces règles. Le Président de la République a annoncé, le 23 novembre 2017, à l'occasion de la clôture du Congrès des maires, son souhait d'améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux. Un chantier est consacré à cette thématique dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. Il pourra se nourrir des travaux engagés par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation qui a constitué un groupe de travail sur le statut des élus locaux et qui devrait présenter ses préconisations d'ici à l'été 2018. Ce sera un élément positif pour engager la recherche d'une solution à la difficulté que vous soulevez. La parole